Cet amendement vise à organiser la publication des déclarations de situation patrimoniale des représentants français au Parlement européen. Actuellement, ces déclarations sont envoyées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, mais ne font l'objet d'aucune publication. constitutionnel, dans sa décision n° 2013-676-DC, avait censuré la publication des déclarations d'élus locaux, il ne s'est pas prononcé sur la publication de celles des représentants au Parlement européen. La publicité se ferait auprès de la préfecture de Paris, dans les mêmes conditions que pour les sénateurs et députés.

Mme la garde des sceaux. Compte tenu de la possibilité offerte aux parlementaires européens en retard de déclaration et de paiement de se mettre en conformité avec leurs obligations fiscales sur invitation expresse de l'administration fiscale, il n'est pas justifié, en cas de manquement persistant, de réduire le champ d'application de la démission d'office aux seuls manquements caractérisés par une particulière gravité. Il n'y a pas lieu non plus de donner au bureau de chaque assemblée un pouvoir d'appréciation du manquement. Au demeurant, la suppression du critère de particulière gravité n'empêchera pas le Conseil d'État d'exercer un contrôle de proportionnalité de la sanction. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons rétablir le dispositif de contrôle juridictionnel et de sanction proposé par le Gouvernement, en l'assortissant d'une sanction d'inéligibilité de trois ans.

de celui que nous mettons en place pour les parlementaires français, il importe que le Conseil d'État, tout comme le Conseil constitutionnel, ait la possibilité de porter une appréciation avant de prononcer

de particulière gravité, nous abaissons ici le niveau de conditionnalité de l'inéligibilité en ne mentionnant que l'appréciation de la

Nous avons introduit dans le projet de loi organique la création d'une dotation de soutien à l'investissement des communes et de leurs groupements ; nous y tenons tout particulièrement, car en aucun cas

améliorer le fonctionnement de la DETR et établir une nouvelle dotation qui, par souci de transparence, ne permettra pas de financer des associations, dont certaines ressemblent parfois fort à des officines politiques, mais à laquelle seront éligibles les tout petits projets d'équipement ou de travaux ruraux qui étaient jusqu'à présent financés

à la création dans la loi organique de la dotation de soutien à l'investissement des communes et de leurs groupements, qui remplira un rôle que la DETR ne pourra jamais remplir. remplir. Cette précision étant apportée, la commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 277

Vous avez la parole

de la République, a toute légitimité à vouloir que les commissions qui attribuent les subventions au titre de la DETR travaillent sous le regard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

Si la confiance n'existe plus, ce qu'exprime l'intitulé, peut-on affirmer que les mesures proposées restitueront la confiance ? Où se situe le seuil entre confiance et défiance ?

Pour moi, il s'agit avant tout d'affirmer une éthique et une exemplarité. Ce mot revêt un sens simple pour tous : « faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, et les lois sont faites pour ça », comme le précise Catherine, une citoyenne qui a apporté une contribution sur la plateforme « Parlement & citoyens » où, avec mon collègue Joël Labbé, nous avons mis en consultation publique ce projet de loi et nos amendements.

d'honnêteté intellectuelle et d'exactitude que la commission a cherché un autre intitulé. Je reconnais que celui que nous avons trouvé est d'une très grande platitude, mais il me semble mieux refléter la réalité de ce texte. Monsieur Doligé,

instaure des régulations qui imposent des comportements à ceux qui n'auraient pas suffisamment de morale pour se les imposer eux-mêmes spontanément. À mon sens, il n'est donc pas approprié de parler de loi de moralisation. C'est du reste ce qu'ont décidé dans un même ensemble le Président de la République,

nos bonnes intentions, n'aura pas atteint totalement son objectif, c'est-à-dire faire savoir que nous oeuvrons tous pour le bien commun, que nous avons une obligation de probité, que nous sommes tenus de lutter contre les conflits d'intérêts,

Le scrutin est ouvert.

Madame la présidente, comme je l'avais annoncé dès la nuit dernière, en application de l'article 43, alinéa 4, du règlement, je demande une seconde délibération de l'article 4 du projet de loi.

peut être renvoyé, sur décision du Sénat, à la commission pour une seconde délibération, à condition que la demande de renvoi ait été formulée ou acceptée par le Gouvernement ou acceptée par le Gouvernement ». Le Gouvernement accepte-t-il cette demande de seconde délibération ? Le Gouvernement l'accepte très favorablement ! Je consulte

lorsqu'il y a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la commission, qui doit présenter un nouveau rapport

de la commission des lois qui a été supprimé la nuit dernière, en y intégrant les amendements qui avaient fait l'objet d'un avis favorable

Le scrutin est ouvert.

Un certain nombre de nos propositions ont été sévèrement frappées par l'application de l'article 45, alinéa 1 de la Constitution sous prétexte qu'elles seraient des cavaliers législatifs.

qui fondent son application, nous n'avons aucune voie de recours. Ce point devra évoluer dans une future réforme de notre règlement : la confiance passe aussi par là Nous n'avons donc pu débattre de dispositions essentielles permettant de retrouver la confiance de nos concitoyens. Je veux bien entendu parler du scrutin proportionnel, du droit d'amendement citoyen, de la reconnaissance du vote blanc, de la généralisation des consultations citoyennes et de bien d'autres choses encore. En revanche, nous avons tout de même pu faire faire évoluer quelques dispositions de notre droit. Nous avons complété la liste des délits entraînant une peine d'inéligibilité quasi automatique, sauf décision spécialement motivée du juge, en y ajoutant le délit d'abus de biens sociaux,

Nous aurions aimé aller plus loin quant aux conditions d'inéligibilité ; nous nous en sommes longuement expliqués, madame la garde des sceaux, y compris par rapport à la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

avancée importante, nous avons décidé que les indemnités de fonction seraient elles aussi fiscalisées

Pour ce qui est des emplois familiaux, après un temps de réflexion, voire d'hésitation, il y a eu un vote magnifique. La très large majorité

loi, pour la première fois, des dispositions relatives aux collaborateurs parlementaires. Grâce à notre travail, à celui de la commission

Il était utile de le faire, en particulier sur les conditions de licenciement ou de rupture. C'est la première fois que cela est fait : c'est une avancée dont nous devons nous réjouir. Pour toutes ces raisons, notre groupe votera ce texte.

Pour en revenir à ce projet de loi, je me félicite que trois de nos amendements ont été adoptés : celui sur le « verrou de Bercy », celui sur la peine complémentaire d'inéligibilité

qui pourraient diminuer les moyens de travail des parlementaires si nous ne sommes pas rigoureux et égalitaires quant à l'utilisation à l'issue du débat, des pans entiers de l'immoralité de notre société ne sont pas pris en compte : le lien entre médias, argent et politique, la question du mode de scrutin et de la représentativité des parlementaires, celle de la dérive monarchique de nos institutions et, bien sûr, la nécessité d'actions contre de détestables pratiques économiques et financières. Ce texte comporte donc des failles qui, de notre point de vue, empêchent de répondre aux vrais enjeux démocratiques qui conditionnent la confiance. En fin de compte, nous ne nous opposerons pas à ce texte, mais nous ne le voterons pas non plus : nous nous abstiendrons.

Le scrutin est ouvert.